Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer en votre nom la présence dans notre tribune d’honneur de Mme Malgorzata Kidawa Blońska, maréchal du Sénat de la République de Pologne, et des trois sénateurs polonais qui l’accompagnent.

aujourd’hui –, occupe de nouveau une place centrale dans le dialogue politique européen. Nos deux pays ont également en commun l’attachement au bicamérisme et au rôle stabilisateur de la Chambre haute. Je me félicite de notre détermination à soutenir ensemble la diplomatie parlementaire, notamment dans le cadre du triangle de Weimar des secondes chambres. Nous recevions d’ailleurs ici même, la semaine dernière, la présidente du Bundesrat.

J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a été publiée. Je rappelle que cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

présentées par MM. Étienne Blanc et Jérôme Durain. La procédure accélérée a été engagée sur ces textes. Il a été décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune. Dans la discussion générale commune, la parole est à M. Étienne Blanc, auteur de la proposition de loi et de la proposition de loi organique. Monsieur

Nous avons écouté et compris ceux dont l’engagement exemplaire – policiers, gendarmes, douaniers, magistrats, greffiers, personnels pénitentiaires – permet à nos institutions de tenir debout. Leur travail constitue notre principal rempart contre les narcotrafics. Nous avons écouté et compris ceux qui travaillent dans les secteurs les plus exposés de nos ports et de nos aéroports. Ils subissent au quotidien la pression des trafiquants. Nous avons écouté et compris nos compatriotes qui vivent à proximité des points de, ceux qui vivent à portée d’une balle perdue, les habitants de ces quartiers gangrénés par le trafic. Nous avons aussi écouté et entendu nos concitoyens d’outre mer, dont les collectivités sont aujourd’hui exploitées par les trafiquants comme zones de rebond, et qui ont parfois le sentiment d’avoir été négligés, voire abandonnés au profit de l’Hexagone. Nous avons aussi entendu le cri de nos élus locaux, notamment de nos maires. Dans toutes les communes de France, des métropoles jusqu’aux villages, ils sont en première ligne face aux trafics. Les travaux de la commission d’enquête ont montré leur remarquable implication. Au cours de nos débats, pensons aux maires de ces petites communes qui se sentent si seuls et si démunis quand un point de apparaît, comme à ceux qui, dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes, jusqu’à présent épargnées par le trafic, se trouvent brutalement confrontés à des règlements de comptes et à des violences inégalées. Après cette nécessaire introduction, j’en viens aux deux propositions de loi qu’il nous revient aujourd’hui d’examiner. Les travaux de la commission d’enquête

et fait vivre environ 240 000 personnes, où l’incarcération ne fait plus peur aux délinquants. Nous avons dressé le portrait d’un pays où les trafiquants utilisent tous les interstices pour pénétrer les institutions et les infrastructures. On peut par exemple se permettre de payer 100 000 euros pour faire déplacer un conteneur dans une enceinte portuaire si les stupéfiants qu’il contient rapportent plusieurs dizaines de millions Nous devons aussi nous souvenir que les trafiquants sont ingénieux. À chaque porte qui se ferme, ils cherchent une fenêtre à ouvrir. Pendant la crise sanitaire de 2020, alors que le confinement limitait les déplacements et, par voie de conséquence, le chiffre d’affaires des trafics, trafics, des systèmes de commandes en ligne avec des livraisons à domicile ont été imaginés. Lorsque nous avons mis en place 100 % de contrôles à Cayenne pour éviter les acheminements par les mules, c’est sur les Antilles que le trafic s’est reporté. Lorsque les grands ports français, celui du Havre notamment, ont pris conscience de la menace, ce sont vers des ports secondaires, notamment des ports de plaisance, que les flux se sont redirigés. La capacité d’adaptation des trafiquants est aussi remarquable en ce qui concerne le blanchiment. Les narcotrafiquants utilisent des moyens aussi nombreux que divers pour dissimuler les fruits de leurs crimes. Ils recourent aux crypto actifs, à des commerces de façade qui font office de blanchisseuses, à des systèmes traditionnels de compensation appelés. Ils s’appuient sur des prête noms pour acquérir des biens immobiliers, des bijoux, des voitures de luxe et même des œuvres d’art qu’ils pourront revendre pour en tirer des liquidités. Parfois même, ils réinjectent leurs fonds dans l’économie légale sans blanchiment préalable, notamment dans les secteurs où les paiements en liquide sont fréquents. Nous le savons, la loi ne pourra pas tout. Des efforts resteront nécessaires hors du périmètre de compétences du Parlement, en particulier sur deux sujets. Le premier sujet, c’est la coopération internationale. Le nombre de délinquants arrêtés et extradés depuis l’étranger demeure trop limité eu égard aux dizaines de criminels du haut du spectre qui continuent à vivre dans le luxe et la tranquillité à Dubaï ou ailleurs, d’où ils poursuivent leurs activités criminelles. Le second sujet, ce sont évidemment les moyens. Je pense aux moyens humains, mais aussi aux moyens techniques et informatiques. Je ne doute pas que le Gouvernement pourra, au cours de cette discussion, nous exposer ses projets pour doter nos services répressifs des outils dont ils ont besoin pour procéder à une lutte efficace. Face à ce constat, que prévoient les deux textes que Jérôme Durain et moi même avons déposés ?

Dans le délai qui m’est imparti, je me concentrerai sur trois mesures. La première mesure, c’est la création du parquet national anti criminalité organisée, le Pnaco. Sa mise en place est urgente au vu de l’état de la menace. Il est essentiel que ce nouvel acteur soit doté de toutes les prérogatives qui lui permettront d’être véritablement un chef de file. Je le dis avec force et en accord avec nos collègues rapporteurs, Muriel Jourda et Jérôme Durain : nous ne devons pas reculer sur les pouvoirs confiés au Pnaco, notamment en matière d’évocation et de coordination, sous peine de créer une immense déception et d’empêcher l’émergence d’un pilotage global à l’échelon judiciaire qui nous fait aujourd’hui défaut. Prenons exemple sur la sagesse de nos prédécesseurs et rappelons nous que le parquet national antiterroriste, dont le principe était pourtant si contesté, est aujourd’hui un éclatant succès. La deuxième mesure concerne la lutte contre le blanchiment. J’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt des échanges qui ont eu lieu au sein de la commission des lois. N’abaissons pas notre niveau d’exigence à cet égard. Demandons à chaque acteur, y compris privé, de prendre sa juste part dans le combat que nous devons mener contre le blanchiment. Alors que nous allons demander des efforts importants à nos concitoyens au vu de l’état dégradé de nos finances, comment comprendraient ils que nous ne menions pas une lutte acharnée contre le blanchiment ? Repérer les fonds suspects dès qu’ils entrent dans le circuit légal, c’est se donner les moyens de les saisir, de les confisquer, donc d’apporter de nouvelles recettes au budget de l’État et au service de la répression de la criminalité. Je vous proposerai d’ailleurs, pour éviter les incertitudes sur l’épineuse question de la prescription, de considérer que ces délits sont toujours occultes, ce qui va permettre de les poursuivre, y compris lorsque des délais importants

C’est pourquoi nous avons limité leur usage à la criminalité organisée et que nous nous sommes attachés à toujours refuser qu’elles puissent être utilisées pour la délinquance de droit commun. C’est également la raison pour laquelle nous avons, pour chacune de ces techniques, prévu des garanties proportionnées à l’atteinte portée à la vie privée : intervention du juge des libertés et de la détention, limitation de la durée de déploiement, exigences sur la motivation de l’usage de telle ou telle technique. Je crois indispensable d’aller encore plus loin dans l’utilisation de ces techniques spéciales. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement afin dans des conditions conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une technique qui permettra d’activer à distance les appareils mobiles, notamment les téléphones. Je vous proposerai de la restreindre aux infractions les plus graves de la criminalité organisée et de prévoir qu’elle ne pourra être déployée que si l’utilisation d’une technique moins intrusive est impossible.

et sans faiblesse. Faisons en sorte que le Sénat soit à l’origine de ce nécessaire sursaut. Les Français nous observent. Ils nous attendent. Il ne faut pas les décevoir. La parole

Bien sûr, toute délinquance est un trouble à l’ordre public, mais le narcotrafic menace véritablement les intérêts de la Nation. C’est pourquoi nous devons nous doter d’outils qui soient à la mesure de ce péril.

Des commerces ouverts sans avoir rien à vendre, mais qui ont pourtant des clients jusqu’au milieu de la nuit ; de très jeunes gens qui sont propriétaires de voitures qui coûtent 200 000 euros, alors que nous ne leur connaissons

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres d’État, mes chers collègues, j’adresse d’emblée mes vifs remerciements aux forces engagées dans la lutte contre la criminalité et réaffirme mon plein soutien aux élus qui subissent les conséquences des trafics.

Soyons à la hauteur de leurs efforts et travaillons, comme eux, avec rigueur et ambition. Il m’appartient, à la suite de Muriel Jourda, d’évoquer deux thèmes majeurs : la procédure pénale et la lutte contre l’emprise du trafic sur notre pays. de loi, relatif à la procédure pénale, est particulièrement dense et technique. Il comporte de nombreuses évolutions indispensables pour que les enquêteurs et les magistrats puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, sans subir le dépassement technologique qui permet aujourd’hui aux réseaux d’échapper à la répression. La proposition de loi prévoit un arsenal complet pour leur faciliter la tâche. Je pense au jugement des crimes commis en bande organisée par des cours d’assises spécialement composées ; à la mise en place de juges spécialisés de l’application des peines, dont nous vous proposerons d’ailleurs de recentrer le périmètre de compétences sur les profils réellement dangereux ; à la création d’un régime exceptionnel d’immunité de poursuites pour les repentis susceptibles de faire tomber un nombre considérable de leurs complices ou de fragiliser les réseaux les plus puissants. enfin à la création d’un statut d’infiltré civil et à la sécurisation des relations entre les policiers et leurs informateurs. Toutes ces évolutions cumulées auront un impact déterminant sur la capacité des services d’enquête à comprendre les réseaux délinquants et à identifier les membres du crime organisé. Gageons que le Gouvernement nous aidera à aller encore plus loin sur ce chapitre en assurant la recevabilité financière de certains amendements utiles pour mettre fin à cette stratégie de la peur grâce à laquelle les trafiquants empêchent les victimes de porter plainte et les témoins de les dénoncer. Le procès verbal distinct

la protection de l’identité des personnes menacées – témoins, infiltrés, informateurs – ou des méthodes d’action les plus sensibles des enquêteurs, lesquelles ne sauraient être révélées sans porter atteinte à la capacité de la police et de la gendarmerie à faire leur travail dans de bonnes conditions. Nous avons constaté, pendant les travaux de la commission d’enquête, que certains outils dont le législateur avait entendu doter les enquêteurs ne pouvaient pas être utilisés, car la description de leur fonctionnement dans le dossier de la procédure viendrait « donner des billes à l’adversaire », comme on nous l’a expliqué : cette situation n’est pas tenable. Nous ne pouvons pas accepter que le contenu de la loi reste platonique. J’espère que nous pourrons nous mettre d’accord sur ce principe et trouver, ensemble, un juste équilibre. Muriel Jourda et moi même avons d’ores et déjà modifié la rédaction de l’article 16 pour y ajouter de nombreuses garanties, essentielles à nos yeux. Ainsi, nous avons prévu le versement au dossier de la procédure de l’ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, qui autorisera le recours au procès verbal distinct. Nous avons également indiqué que le recours à ce procédé devait être nécessaire à la manifestation de la vérité, ce qui impliquera un effort particulier de motivation en amont de tout déploiement. Nous avons par ailleurs précisé les conditions du contrôle de la chambre de l’instruction, dont je rappelle qu’il sera systématique

Les notions de « manœuvre » et de « négligence » risquent de nous faire passer à côté de notre but, puisqu’elles peuvent elles mêmes donner lieu à des contentieux. C’est pourquoi Muriel Jourda et moi même proposerons une réécriture permettant de modifier des dispositions qui sont aujourd’hui le support des stratagèmes dénoncés par la commission d’enquête. c’est une solution plus modeste, mais elle est vraisemblablement plus efficace. Enfin, le titre VI de la proposition de loi permet de lutter contre l’emprise de la criminalité organisée sur nos infrastructures, dans les prisons et dans certains quartiers. La corruption est une gangrène, une arme de choix grâce à laquelle les trafiquants font progresser leur influence délétère dans tout le corps social. L’article 22 viendra garantir une meilleure prévention et une détection plus facile de la corruption, sans stigmatisation. La commission vous proposera un amendement visant à étoffer notre dispositif de détection de la corruption dans les ports, infrastructures éminemment stratégiques pour les narcotrafiquants, un recours renforcé à la vidéosurveillance des installations sensibles. Ce qui nourrit la corruption, c’est parfois l’appât du gain, mais c’est surtout la peur des représailles en cas de refus. Il faut rétablir la confiance dans l’État, dans la protection qu’il peut apporter à ceux qui veulent dénoncer les promesses ou les pressions dont ils font l’objet. De nombreux amendements ayant pour objet les enjeux pénitentiaires ont été déposés : c’est le signe d’une prise de conscience importante et bienvenue. Là encore, l’intervention du Gouvernement pour permettre l’examen d’amendements judicieux, mais qui créent de toute évidence de nouvelles charges financières, sera appréciée sur toutes les travées. conclusion, je rappelle que c’est le Sénat qui, le premier, s’est saisi du sujet du narcotrafic dans son ensemble, en ayant la volonté de trouver des solutions pour que nos institutions reprennent l’ascendant face aux trafiquants. L’exemple de nos voisins montre qu’il ne faut pas prendre le risque d’être dépassé par la menace. N’attendons pas qu’il soit trop tard avant de réagir.

Ce parquet national doit d’abord coordonner l’action de notre pays, notamment l’action publique en matière de lutte contre les stupéfiants et la criminalité organisée.

mais aussi un manquement à la protection que nous devons aux agents de la pénitentiaire, pour qui j’ai évidemment une pensée émue aujourd’hui à cette tribune, à leurs familles et à l’ensemble de la société.

Sur le haut du spectre, l’armature de l’État est beaucoup trop éclatée face à des réseaux et des organisations qui sont parfaitement coordonnées et pilotées. Pour gagner un combat, et plus encore une guerre, il faut des chefs de guerre.

En miroir de cette organisation juridictionnelle, il faut une organisation opérationnelle dans le périmètre qui est le mien, celui du renseignement,

des affaires de criminalité organisée, associer l’ensemble des services de façon très interministérielle. J’y reviendrai lorsque nous débattrons de l’article 1, sur lequel un certain nombre d’amendements ont été déposés. Ils sont importants, mais je suis très attaché à ce que nous

Si on laisse libre cours à la corruption, dans le privé comme dans le public, dans tous les métiers, nos institutions en subiront les conséquences.

C’est aussi une question de crédibilité vis à vis de nos partenaires européens et internationaux que de mieux gérer nos ressources. Par conséquent, notre main ne doit pas trembler face à ces criminels et à leurs trafics. Un travail considérable est accompli chaque jour par les services de Bercy dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, la criminalité organisée, le blanchiment et les flux financiers illicites.

Grâce à son positionnement privilégié en matière de surveillance et de sécurisation des frontières extérieures de l’Union européenne, à l’instar des autres douanes européennes, la douane est à l’origine de 60 % à 75 % des saisies de 60 % à 75 % des saisies de stupéfiants, toutes administrations confondues. Elle collabore avec les services de police judiciaire et avec l’autorité judiciaire ; elle inscrit son action en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le cadre interministériel du plan national de lutte contre les stupéfiants. Tracfin, lui, est capable d’identifier les avoirs criminels des têtes de réseau du narcotrafic, que ces avoirs soient situés en France ou à l’étranger, et il peut organiser la saisie rapide de leurs comptes bancaires en France et révéler les activités économiques des groupes criminels.

nos services ont permis de mettre au jour des réseaux structurés agissant bien au delà des frontières françaises, ce qui a facilité le travail des magistrats.

nous rassemble autour de son ambition et de ses objectifs, car il s’agit bien d’une priorité nationale. Ce texte constitue une étape majeure pour donner à nos services respectifs, chacun dans son champ de compétence, les outils et les moyens de leur action, dans un contexte où les criminels, eux, font preuve à tous égards d’une grande ingénierie, d’une grande agilité, et disposent de moyens matériels et financiers inédits. Je veux être claire, nous ne pouvons prendre aucun retard par rapport aux trafiquants. L’État doit pouvoir les traquer partout où ils sévissent.

pour bloquer l’accès aux financements en complément de l’action judiciaire, dans les cas de fuite ou pour élargir les actions aux personnes de l’entourage et aux sociétés écrans.

Ces avancées sont précieuses pour les services concernés, mais nous souhaitons aller encore plus loin. Ah… Lors des débats, nous vous proposerons plusieurs amendements visant à renforcer la répression du blanchiment et à entraver davantage encore l’action des criminels.

C’est le sens des dispositions que nous vous présenterons, permettant notamment aux agents de la douane d’avoir accès aux données de certains opérateurs privés dans les secteurs des transports et de la logistique.

Cette extension permettra, pour la première fois, à ce service de traiter des informations émanant de personnes physiques. Elle permettra aux lanceurs d’alerte de signaler tout type de faits, notamment des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants. Les flux financiers sont également au cœur des enjeux de la lutte contre les trafics. L’extension de la présomption de blanchiment douanier, notamment aux crypto actifs, permettra d’inverser la charge de la preuve de la provenance délictueuse des fonds : ce sera aux fraudeurs

ou le matériel issu des trafics, mais aussi d’entraver la circulation des flux financiers massifs générés par ces trafics. La création de la procédure d’appréhension des comptes bancaires et des instruments financiers en cas de notification d’infractions douanières

Par ailleurs, l’ancienne ministre de la fonction publique que je suis note avec une grande satisfaction que les agents des douanes pourront se pseudonymiser. protéger pleinement face aux trafiquants qui, eux, ne connaissent pas de limites. Je salue aussi la possibilité que vous souhaitez offrir aux enquêteurs de l’Onaf de faciliter leur saisine en matière de blanchiment du produit des infractions à la législation des stupéfiants, qui lui permettra d’être encore pleinement vous le voyez, il est urgent d’agir. Le Gouvernement n’a pas qu’une vision régalienne des sujets et inclut pleinement les enjeux financiers. L’État sera fort, grâce à vous, et je vous en remercie.

mes chers collègues, nous connaissons les conséquences humaines et sociales dramatiques du narcotrafic dans la quasi totalité des territoires de la République. Nombreux sont les quartiers qui portent les stigmates d’un trafic à ciel ouvert.

Ce que nous pouvions considérer il y a quelques années comme des faits divers, des épiphénomènes individuels, est devenu un fait social pour notre nation entière.

Les trafiquants ont développé des réseaux très organisés. Cette expansion s’accompagne d’une augmentation alarmante de la violence, ainsi que de faits de corruption très préoccupants. Certains territoires d’outre mer sont particulièrement vulnérables. Leur géographie, stratégique, en fait des plaques tournantes du trafic de cocaïne et de cannabis. Les rapporteurs l’ont souligné : nous observons également une véritable ubérisation du trafic, allant jusqu’à la création de centres d’appels pour assurer des livraisons à domicile. Les criminels rivalisent d’ingéniosité pour contourner la répression. Cette sophistication des méthodes conduit à ce que le trafic se structure comme une industrie, à l’échelon tant national qu’international.

l’organisation d’une lutte efficace contre le trafic ne nous exemptera pas d’un débat de société sur les drogues, sur les explications sociales de l’addiction, pour comprendre comment des jeunes oubliés des politiques de la ville tombent aujourd’hui dans les mains des trafiquants.

: la réponse sécuritaire et pénale. Le consensus sénatorial est attendu par nos concitoyens. Je ne ferai pas l’inventaire des dispositifs

C’est une très bonne chose, car il y a une dimension tentaculaire dans le narcotrafic, qui s’accomplit suivant des procédés innombrables. Il ne faut pas nous restreindre ! Nous saluons également l’ensemble des dispositifs proposés en vue d’endiguer le blanchiment d’argent. D’autres outils d’ordre procédural pourraient également voir le jour. Je pense à la création de dossiers coffres ou au recours au procès verbal distinct pour protéger les techniques d’enquête sensibles. Il s’agit indéniablement d’une atteinte au principe du contradictoire, constituant un pilier du procès équitable. je vous invite à veiller à ne pas fragiliser les droits de la défense. La délibération parlementaire que nous nous apprêtons à avoir est importante pour trouver des solutions de compromis qui garantissent la protection des droits et des libertés tout en maintenant un exigeant niveau d’efficacité. À mon sens, la mesure est suffisamment encadrée, limitée et proportionnée à l’objectif qu’elle vise. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, tout en espérant que ce texte soit accompagné des moyens financiers nécessaires,

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic prolonge opportunément le travail accompli par la commission d’enquête sénatoriale, qui était présidée par Jérôme Durain et dont le

La France reste un pays sûr. Nous avons un État qui fonctionne. Notre police et notre justice agissent. Nous devons leur permettre de s’adapter, car nous entrons dans une nouvelle ère. L’Amérique latine, avec 8 % de la population mondiale, totalise 37 % des homicides. Plus des deux tiers de ces meurtres sont attribuables à des groupes criminels. Traditionnellement, les cartels contrôlaient des territoires limités et se spécialisaient dans un seul produit, généralement la cocaïne. Aujourd’hui, ils s’internationalisent et se diversifient rapidement. Ils s’impliquent de plus en plus dans le trafic d’êtres humains et de produits illégaux, dans les kidnappings et l’extorsion.

Étienne Blanc l’a bien dit : nous pouvons voter toutes les lois du monde, si nous ne mettons pas les moyens en face, les résultats ne seront pas au rendez vous. Pays producteurs et pays consommateurs ne peuvent se renvoyer la balle. Ils sont les deux faces de la même pièce.

Nous y avons découvert des sacs de précurseurs chimiques fabriqués en Chine, qui entrent à 60 % dans la composition de la cocaïne. Ces précurseurs chimiques peuvent être commandés sur internet. Ils composent également les drogues de synthèse comme le Fentanyl. Un vendeur de Fentanyl dans les rues de New York gagne 30 000 dollars par semaine. Les États Unis sont passés de quelques centaines de décès liés à ce produit au début des années 2010, à plus de 70 000 en 2021, pour franchir la barre des 120 000 décès en 2023. Cette année là, le président Biden a ajouté la Chine à la liste américaine des principaux pays producteurs de drogues illicites au monde. Les mafias chinoises assurent le blanchiment de ces profits au travers de casinos, d’immobilier et de sociétés écrans diverses. Comme notre commission d’enquête l’a révélé, Hong Kong est devenu le trou noir du blanchiment. Si louables que soient les avancées proposées dans ce texte, que le groupe Union Centriste soutiendra, nous sommes conscients que le volet répressif ne résoudra rien à lui seul. Le premier décès officiel par overdose enregistré en France date de 1969. Nous en comptons actuellement plusieurs centaines par an. Sur les routes, un décès sur cinq implique un conducteur ayant consommé de la drogue. Au delà des mesures d’urgence proposées dans ce texte, sur lesquelles reviendra Pascal Martin, il nous faudra des politiques beaucoup plus élaborées sur le long terme, avec des efforts importants pour la prévention, en particulier en faveur de pour enrayer la violence liée à la drogue tout en préservant nos libertés publiques. La guerre contre le narcotrafic est mondiale. Pour la gagner, il faut adopter une approche européenne, en donnant de véritables moyens à la coopération internationale contre le crime organisé

C’est d’ailleurs ce qui m’a poussé, avec mes collègues Marie Arlette Carlotti et Guy Benarroche, à demander au président Larcher la mise en place d’une commission d’enquête sur le narcotrafic. Enfant des quartiers nord de Marseille, je sais pourtant que ma ville, mes quartiers, ne se résument pas à cela – tant s’en faut. Pourtant, comment ne pas voir la progression continue des trafics, de plus en plus organisés, structurés et, j’ose le mot, de mafias structurant ces trafics ?

pays. Oui, cette problématique est bien une problématique nationale, et même internationale. Je voudrais ici rendre hommage au député communiste italien Pio La Torre, assassiné par la mafia en 1982 après avoir mené une vie de combat contre ces organisations criminelles. rendre hommage aussi à François Billoux, député communiste de Marseille, ministre, qui, dès 1936, lançait une grande campagne intitulée « Marseille propre », pour lutter contre les mafias de l’époque. Le communiste que je suis sera toujours pour la lutte acharnée contre ces réseaux et ces mafias. Certaines mauvaises langues mal intentionnées pourraient trouver contre intuitif qu’un communiste appelle à l’ordre. Ce n’est pas du tout ce que les premières victimes de ces mafias sont bel et bien les personnes les plus fragilisées, les plus vulnérables et les plus précaires. Ce sont leurs quartiers, leurs maisons, leurs familles qui sont exploités par les bandes mafieuses. Si l’État les a abandonnés, les trafiquants, eux, se montrent bien présents, gangrenant notre pays et profitant des failles de notre État social. Si je salue ici le travail de mes collègues sur cette proposition de loi, il nous faudra aussi réinvestir tous les territoires de la République. Là où l’État est fort, le narcotrafic recule. Là où l’État est faible, les mafias prospèrent.

Nombreux sont ceux qui tirent la sonnette d’alarme face à cet abandon. Il faut protéger aussi tous les professionnels particulièrement exposés aux narcotrafiquants, plutôt que les présumer coupables ou complices. Je pense bien sûr aux avocats, au personnel des ports, aux dockers, aux agents pénitentiaires ou encore aux douaniers. C’est parce qu’ils sont en première ligne face aux réseaux de narcotrafiquants qu’il nous faut assurer leur protection. Nous avons déposé plusieurs amendements en ce sens. Enfin, il nous faut agir avec cohérence et détermination à chaque étape de la lutte contre le narcotrafic.

contre la criminalité organisée. Nous attendons donc le retour de la police judiciaire, seule apte à faire face à la criminalité organisée. La cohérence et la détermination à chaque étape de la lutte contre le narcotrafic doivent aussi s’incarner dans nos relations diplomatiques. La France doit davantage hausser le ton contre les pays producteurs de drogues, que ce soit le cannabis, la cocaïne ou l’héroïne. S’attaquer aux mafias, c’est aussi s’attaquer aux lieux de production qui prospèrent à travers le monde, parfois même, malheureusement, avec la complicité de certains États. Par conséquent, malgré les mises en garde émises et notre vigilance lors de l’examen du texte, notre groupe, convaincu que la lutte contre le narcotrafic s’intègre dans un projet de développement économique, social, démocratique et populaire, et dans un souci de responsabilité,

Nous regrettons l’absence de mesures d’information pour éviter l’entrée dans la consommation, sur les parcours de soins, sur la prise en charge des addictions, sur l’intérêt de légaliser ou de dépénaliser certains usages : aucune politique de santé publique, Rien non plus sur le volet économique et social, levier majeur de la lutte contre le narcotrafic. Rien sur la politique de la ville. Rien sur la lutte contre la précarité. Rien sur le logement, sur l’insertion par l’école et par le travail.

de moyens, celles ci ne permettront pas de déjouer le piège du narcotrafic. Les nombreuses solutions avancées seront déterminantes dans les domaines judiciaire, policier, administratif et financier, sur le blanchiment et la corruption. La plupart des mesures proposées vont dans la bonne direction et sont, je le répète, indispensables. Le narcotrafic est le du capitalisme libéral mondialisé. Il ne se limite pas aux stupéfiants. C’est un système de criminalité organisée, qui a comme composante principale et native le trafic de drogues. Nous apprécions que le texte sorte de la focalisation sur le bas de la chaîne, les produits stupéfiants, le consommateur, pour enfin viser plus loin, frapper les trafiquants au porte monnaie s’attaquer à un système globalisé. Les articles sur le blanchiment étaient attendus, ils sont bienvenus. Nous saluons la nécessaire prise en compte de la corruption, phénomène qui était très nettement sous évalué par toutes les administrations Nous resterons toutefois très vigilants quant à l’équilibre du texte. Ainsi, nous examinerons comment sera améliorée la chaîne du traitement judiciaire et policier du narcotrafic. Notre combat acharné et déterminé contre ce fléau ne doit pas s’effectuer au détriment des droits de l’ensemble des justiciables et de la défense.

Loin des caricatures, nous souhaitons mettre fin à la délinquance liée au trafic et à une criminalité qui blesse, tue, rackette, terrorise nos villes, essaie de corrompre les plus précaires et constitue un danger pour la sûreté et la tranquillité publiques ! Le narcotrafic atteint toutes les sphères et tous les domaines de notre société.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis pour modifier notre arsenal juridique, afin de lutter contre un mal qui fait des ravages partout en France, dans nos moyennes et grandes villes, nos campagnes, sans oublier nos territoires ultramarins le trafic de stupéfiants. Je tiens à saluer l’excellent travail de Jérôme Durain et d’Étienne Blanc au sein de la commission d’enquête, puis dans la rédaction de ce texte. Celui ci a vocation à poser les premiers jalons d’un État plus fort et mieux armé dans la lutte contre le narcotrafic, mais aussi, et surtout, contre la violence exacerbée que celui faisant de nombreuses victimes, souvent très jeunes. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain salue d’abord la réorganisation indispensable des acteurs de cette lutte, qui ont besoin d’une véritable spécialisation. Cela passe par le renforcement de l’Office anti stupéfiants par la création d’un parquet national anti criminalité organisée, avec une meilleure coopération et une coordination avec les juridictions interrégionales spécialisées. Nous nous félicitons également des nouveaux outils visant à lutter contre le blanchiment, comme la procédure d’injonction pour richesse inexpliquée ou le gel judiciaire des avoirs. En effet, « frapper au portefeuille » les trafiquants semble devenu parfois beaucoup plus dissuasif que la menace

Je l’ai souligné, ce texte pose les premiers jalons. Soyons clairs : si nous sommes désarmés face au narcotrafic, c’est parce que nous n’avons pas les moyens financiers de lutter contre. Notre pays fait partie des pays européens qui investissent le moins dans leur justice. Nous devons investir massivement dans toute la chaîne pénale pour recruter des magistrats et des fonctionnaires de justice capables de faire face à une prolifération d’affaires. ce n’est pas parce que notre justice manque cruellement de moyens qu’il faut désarmer les avocats en violant les droits de la défense. Nous refusons de remettre en cause la probité des avocats qui ne font qu’utiliser les voies de droit légales existantes, afin d’assurer la défense de leurs clients. Le code de procédure pénale est un élément constitutif clé de notre État de droit. Les plus grandes précautions s’imposent quand il s’agit d’y toucher.

et de nos libertés individuelles. Nous vous proposerons des amendements en ce sens. Enfin, nous saluons les dispositifs visant à lutter contre la pénétration du narcotrafic en prison. Au travers de nos amendements, nous restons fidèles à nos demandes constantes relatives au respect des conditions de détention dignes, élément primordial, notamment afin de lutter contre la récidive.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres d’État, mes chers collègues, le 11 septembre 2023, Socayna, 24 ans, était tuée chez elle par la balle perdue d’un narcoterroriste. Elle habitait non pas dans la banlieue de Bogota ou de Mexico, mais dans une résidence du dixième arrondissement de Marseille. Cette tragédie a suscité émotion et colère à travers tout le pays, et puis… on est passé à autre chose ! Faut il attendre que des policiers ou des magistrats soient tués ? Faudra t il que le ministre de la justice soit menacé d’enlèvement, comme c’est le cas en Belgique, pour que vous agissiez, afin d’éviter que la France ne devienne à son tour un narco État ? Ce terrorisme du quotidien entraîne l’incarcération d’habitants de résidences et de cités entières chez eux, soumis aux contrôles aux frontières des territoires conquis, où les agents des services publics, pompiers et médecins compris, sont, comme je l’ai été moi même, arrêtés, contrôlés, et dont le véhicule est fouillé. Les plus libres de nos compatriotes qui vivent ce terrorisme de moyenne ampleur ont honte d’inviter leurs proches chez eux, car il leur faudrait passer le contrôle des choufs. Oui, ils ont honte d’habiter dans certains quartiers de la deuxième ville de France ! Dans ce contexte, trouver un avec les dealers et légaliser le cannabis, comme le souhaite le maire gauchiste de Grenoble, reviendrait à officialiser la victoire de ce terrorisme. C’est sur les épaules de ces politiques gauchos collabos que la honte devrait lourdement reposer ! Parlons en, des collabos ! De plus, 50 % des petites mains du trafic interpellées par la police à Marseille sont des clandestins. Eh oui, monsieur le ministre de la justice, cette submersion est non pas un « sentiment », mais une réalité ! D’ailleurs, les appellations, Wakanda et DZ Mafia – DZ pour Algérie –, évoquent des systèmes de valeurs explicitement étrangers. Pourtant, pas une fois, vous n’avez prononcé le mot « immigration » lors de votre venue à Marseille, monsieur le ministre de l’intérieur. Pas une fois il n’y aura pas de lutte efficace contre le narcoterrorisme sans lutte déterminée contre l’immigration. Vous avez ignoré mon témoignage d’élu de terrain, que je livre depuis dix ans dans cet hémicycle et depuis vingt ans à Marseille Entendez l’appel des victimes de ce trafic, en instaurant une prévention tous azimuts, car la drogue c’est aussi et d’abord une affaire de santé publique, et en rétablissant chaque maillon de la chaîne répressive contre le narcotrafic. narcotrafic. Du producteur au consommateur, la lutte doit être impitoyable. En amont, pour les pays producteurs, il faut une trumpisation de nos mesures ! Pas de coopération ? Plus de visas ! Plus d’aide au développement ! Plus d’étudiants ! En aval, verbaliser lourdement les consommateurs avec saisies sur salaire ou prestations sociales, sortie de Schengen, expulsion de tous les clandestins et déclaration d’un état d’urgence avec l’appui de l’armée dans les territoires conquis ! Et que l’on ne vienne pas me bassiner avec la pseudo raison sociale du trafic. Il n’y a pas de trafic de drogue en Corrèze ou dans la Creuse, les deux départements les plus pauvres de France,… N’importe quoi ! Il faut bénéficient de la politique de la ville et de son torrent d’argent public depuis des décennies ! C’est fini ! Alors que les magistrats marseillais craignent le financement des campagnes électorales par des organisations narcoterroristes,… Il faut conclure, mon tout nous démontre que les narcoterroristes sont déterminés à nous faire la guerre. Fini ! Non seulement il faut faire la guerre aux narcoterroristes, mais il faut avant tout se doter des moyens de la gagner

Trop longtemps, trop souvent, les stupéfiants ont été considérés sous le seul angle de l’usage récréatif ou des drogues douces. Force est de constater que ni notre arsenal législatif ni notre politique pénale n’ont permis de faire reculer la consommation ou d’endiguer les trafics. À l’heure actuelle, les stupéfiants sont en France un marché juteux, qui pèse entre 3 milliards d’euros En 2024, les quantités de drogue saisies par les autorités progressent : 47 tonnes de cocaïne, 88 tonnes de cannabis. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige Ils sont le reflet, mes chers collègues, des névroses de notre société. Ville, banlieue, campagne – ne vous en déplaise, mon cher collègue –, la drogue est désormais partout dans notre pays. Plus d’un million de nos concitoyens ont ainsi consommé de la cocaïne en 2023. Derrière les récréations de certains, derrière la consommation personnelle, il y a aussi les victimes abattues par les trafiquants de drogue et les tenants d’autres trafics. Les consommateurs de notre pays détournent sans doute les yeux des crimes atroces commis par les cartels latino américains. Pourtant, comme l’a si bien décrit le si courageux Roberto Saviano, la violence est consubstantielle au trafic de drogue. À mesure que les stupéfiants affluent sur le territoire, le nombre de morts augmente. Sans compter les décès liés à la consommation de drogue, quatre vingts personnes ont ainsi été tuées par les réseaux mafieux en 2023. La drogue ne tue pas seulement les trafiquants ou les usagers. Elle menace parfois la vie de Français qui n’ont aucun lien avec ce commerce. Ce fut le cas encore une fois à Grenoble d’une adolescente de 16 ans blessée par balle le 4 janvier dernier. Beaucoup n’ont pas la chance d’en réchapper. Un conducteur de VTC qui refusait d’acheminer un petit tueur à gages de 14 ans vers sa cible a été abattu par son jeune client. Une jeune femme de 24 ans, atteinte par une balle perdue d’une arme de guerre, est morte dans sa chambre à Marseille. Ces victimes doivent peser sur la conscience des consommateurs de drogue. Ce sont eux qui financent et arment les trafiquants. Si nous entendons mettre un réel coup d’arrêt au développement des trafics, si nous entendons protéger nos concitoyens de ces réseaux, il nous faudra aborder ce sujet. Hélas, la consommation de drogue ne fait pas partie du périmètre de ce texte. C’est sans doute pour ne pas disperser les efforts du Sénat, sans doute aussi parce que nous n’avons pas les mêmes opinions en la matière. Nous sommes assez navrés d’entendre certains nous expliquer que le trafic de stupéfiants est seulement une conséquence du capitalisme et du libéralisme, surtout lorsque ce sont précisément ceux qui prônent la légalisation – celle ci ne semble pas vraiment avoir fait ses preuves dans les pays où elle est en vigueur – et qui imaginent que l’on lutte contre la criminalité à coups d’aides sociales. Ce n’est pas notre vision. Il est affligeant d’entendre dire que la pauvreté conduit automatiquement à la délinquance. En plus d’être clairement faux, cela revient à bafouer ceux de nos concitoyens qui gagnent leur vie en travaillant honnêtement À l’heure où tous nos territoires sont affectés par les trafics, le vent tourne. Je ne doute pas que nous serons nombreux à voter finalement en faveur de cette proposition de loi. La commission d’enquête sénatoriale, à l’origine de ce texte, a démontré la nécessité de spécialiser la chaîne pénale chargée de traiter les affaires de criminalités organisées. Cette matière, comme les affaires de terrorisme ou encore les affaires financières, présente une particulière complexité et menace gravement notre société. La proposition de loi modernise et améliore également la procédure applicable à la poursuite des trafics dans le cyberespace. Les trafics prolifèrent de manière exponentielle grâce aux nouvelles technologies, qui deviennent le premier vecteur du crime organisé et des trafics en tous genres. Il faut que cela cesse.

nous examinons aujourd’hui une proposition de loi nécessaire pour sortir notre pays du piège du narcotrafic. Son corollaire est une proposition organique fixant le statut du procureur national anti stupéfiants. Face à la progression incontrôlée du phénomène en question, nous, parlementaires, devons apporter une réponse claire, sans compromissions ni ambiguïtés. Ces textes ambitieux sont le fruit du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France, sur l’initiative du groupe LR. Ce rapport transpartisan, adopté à l’unanimité le 14 mai dernier, fait le constat froid et sans appel de la situation critique que connaît notre pays. Les textes déposés par nos collègues les sénateurs Étienne Blanc et Jérôme Durain Durain transposent et mettent en œuvre à l’échelon législatif les recommandations de la commission d’enquête. Le narcotrafic se développe aujourd’hui largement sur le sol national, notamment dans les villes moyennes, mais aussi dans les zones rurales, autrefois épargnées. Il est très fortement présent dans mon département, les Pyrénées Orientales, notamment en raison de la position frontalière de celui ci avec l’Espagne. En effet, les axes routiers structurants, comme l’autoroute A9, sont très empruntés par les trafiquants, acheminant les stupéfiants provenant du Maroc, d’Afrique et des Antilles. Ainsi, en 2024, les forces de l’ordre ont saisi 18 tonnes de résine et d’herbes de cannabis, 495 kilogrammes de cocaïne et 215 grammes d’héroïne. Par rapport à 2023, les saisies de drogues dures ont explosé. À titre d’exemple, le point de le plus important situé à Perpignan produit à lui seul entre 35 000 euros et 50 000 euros par jour de chiffre d’affaires. Ces revenus sont aujourd’hui gérés depuis l’étranger ; nous y reviendrons dans la discussion des articles. Par ailleurs, si les convois de type sont toujours d’actualité, l’activité des trafiquants s’inscrit désormais dans un schéma de type « rouleurs stockeurs » spécialisé dans le convoyage de stupéfiants entre l’Espagne et la France. Le département des Pyrénées Orientales est aujourd’hui une place logistique de premier ordre pour le narcotrafic. C’est devenu une véritable problématique du quotidien pour l’État et les collectivités territoriales. Je souhaite d’ailleurs insister sur quelques préoccupations majeures de nos acteurs de terrain, les élus locaux, les magistrats et les policiers, trop souvent confrontés à ce fléau. Tout d’abord, les établissements de type épiceries de nuit posent un véritable problème. En effet, ils servent très souvent de façade au trafic de stupéfiants, causant ainsi de graves troubles à l’ordre public. Les élus sont confrontés quotidiennement à la difficulté de freiner l’implantation de ces commerces ou de les fermer. Désormais, de nombreux maires sont la cible d’agressions par ces pseudo commerçants. C’est pourquoi je n’ai pas manqué de soutenir l’amendement des rapporteurs tendant à prolonger le délai de fermeture administrative des commerces prononcée par le préfet. Cette mesure est fortement attendue dans nos territoires. Le parc locatif public est une cible privilégiée pour les narcotrafiquants. Un certain nombre de dispositions portent sur le sujet. Les bailleurs sociaux sont aujourd’hui totalement dépourvus de moyens légaux efficaces face à l’ampleur des trafics. C’est dans cet esprit que j’ai demandé, en accord avec le Gouvernement, la rédaction à terme d’un Enfin, l’assassinat des deux agents à Incarville – cela a été évoqué tout à l’heure, notamment par M. le garde des sceaux –, lors de l’évasion de Mohamed Amra, dit La Mouche, a rappelé que la sécurisation des convois pénitentiaires circulant sur la voie publique était un sujet majeur. En effet, les équipages de ces convois sont exposés à de graves dangers du fait de réseaux de criminalité organisée ne reculant désormais devant aucun moyen pour permettre l’évasion ou atteindre une personne détenue au cours de son transport. Les agents de l’administration pénitentiaire m’ont fait part de leurs craintes, pour ne pas dire de leurs peurs, désormais d’assurer ces convois. Ils demandent notamment la mise en place de tribunaux délocalisés et la tenue d’audience en visioconférence. Il est de la responsabilité de l’État de mettre en œuvre tous les moyens pour protéger ces hommes et ces femmes de tous les risques d’actions violentes. C’est dans cet esprit que j’ai déposé un amendement visant à doter l’administration pénitentiaire d’outils efficaces de surveillance et de protection. Ainsi, les caméras embarquées à bord des véhicules permettront de procéder à la captation d’images pendant les opérations de transport des personnes détenues, facilitant le recueil de preuves aux fins de judiciarisation des incidents survenus sur la voie publique et la poursuite de leurs auteurs. Aujourd’hui, nous sommes à un véritable point de bascule. Le piège du narcotrafic se referme lentement sur notre pays. Nous devons agir de toute urgence. Bien que nos ministres aient pris désormais leurs responsabilités face à la gravité de la situation, nous avons nous avons besoin d’outils opérationnels et adaptés dans le cadre de cette lutte. Nous avons déjà pris beaucoup trop de retard face à l’inadaptation de nos droits et les failles de notre système juridique. Nos concitoyens, les forces de sécurité, les acteurs de justice et les élus attendent de la discussion parlementaire que nous menons aujourd’hui des réponses fortes pour sortir de ce piège. Je suis convaincue que nous saurons les leur donner. Pour toutes ces raisons,

Enfin, la France se donne les moyens de lutter efficacement contre le narcotrafic ! Le texte dont nous commençons l’examen entend donner aux autorités françaises les moyens de sortir la France du piège du narcotrafic. Cependant, cette problématique n’est pas nouvelle. le Sénat a publié plusieurs rapports d’informations qui s’évertuaient à chercher des pistes pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Le phénomène a pourtant explosé au cours de ces dernières années. J’en veux pour preuve l’augmentation des saisies de cocaïne : de 27 tonnes en 2022, nous sommes passés à 47 tonnes l’an passé. Loin de moi l’envie de juger le travail de mes prédécesseurs, mais nous devons avoir la maturité nécessaire pour admettre qu’à chaque fois la problématique avait été appréhendée des thématiques spécifiques.

Je ne peux que féliciter mes collègues Jérôme Durain et Étienne Blanc, respectivement président et rapporteur. Je suis d’ailleurs extrêmement flattée d’avoir contribué à cette entreprise. Jamais nous n’avons eu une vision aussi globale du narcotrafic sur l’ensemble du territoire français. Jamais les outils et les armes nécessaires pour mener à bien cette lutte n’avaient été aussi clairement répertoriés. Ce texte renforce à la fois le volet pénal, consolide les moyens pour lutter contre le blanchiment de capitaux et crée un parquet national spécialisé, afin d’incarner la figure unique de la poursuite et de la répression de la criminalité organisée. En tant que Guyanaise, je tiens à rappeler que nos territoires ultramarins subissent de plein fouet ce trafic de stupéfiants à cause de leur proximité avec les pays producteurs. C’est en 2010 que ce trafic a été mis en lumière de manière significative en Guyane. Ce fléau n’a épargné aucune famille guyanaise, s’enracinant dans les quartiers dans lesquels se mêlent pauvreté et manque d’opportunités professionnelles. Par la suite, le phénomène s’est amplifié en Martinique et en Guadeloupe quand le passage à l’aéroport de Guyane est devenu plus complexe. Par conséquent, je me félicite qu’une partie du texte y soit consacrée. Il est proposé de prolonger la garde à vue médicale et de renforcer les peines d’interdiction d’embarquer dans nos territoires ultramarins pour enrayer le phénomène des « mules ». Nous devons à tout prix protéger notre jeunesse. Justement, c’est là que le bât blesse. Le texte, aussi riche soit il, fait peu de cas de notre jeunesse. La mère de famille et ancienne maire que je suis ne peut pas accepter que la lutte contre le trafic de stupéfiants ne soit qu’une question de répression. Elle doit aussi être une question de prévention, de solidarité et d’accompagnement. Il ne s’agit pas uniquement de démanteler les têtes de réseau, il faut aussi offrir des alternatives aux jeunes, qui, faute de choix, se laissent entraîner dans cette spirale infernale. Le rapport sénatorial d’information de 2020 sur le trafic de stupéfiants en provenance de la Guyane suggère avec force le développement de l’offre de formation pour les jeunes. Il a aussi été question du renforcement de la prévention auprès des jeunes, les cibles privilégiées des commanditaires. Ces recommandations n’ont jamais été suivies d’effets ; je le regrette amèrement. Nous devons plus que jamais privilégier une approche humaine et globale. Par ailleurs, je constate avec satisfaction la mise en œuvre de la compétence universelle en matière de trafic de stupéfiants. La Marine nationale, surtout dans les Antilles, pourra plus facilement intervenir en haute mer pour contrôler les navires soupçonnés de participer à un trafic sur notre sol. Je note toutefois que la commission, par volonté de respecter le droit international, a encadré ces opérations. Enfin, je regrette que l’idée de renforcer la coopération avec les pays producteurs de cocaïne n’ait pas pu être transposée dans ce texte, alors qu’elle figure clairement dans le rapport de la commission d’enquête. Avant de conclure, je tiens une nouvelle fois à saluer le travail de la commission d’enquête et de nos rapporteurs ici présents. Cette proposition de loi demeure très ambitieuse et va dans le bon sens. La France se dote enfin de moyens pour importuner les réseaux qui gangrènent nos villes et favorisent l’insécurité. Pour ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. La parole

la commission d’enquête du Sénat a terminé ses travaux par un constat sans appel : aujourd’hui, le narcotrafic constitue une menace pour les intérêts fondamentaux de notre nation. Nous sommes face à un point de rupture. Nous pouvons peut être encore redresser la barre sans basculer, comme certains de nos voisins européens, dans une véritable mexicanisation de notre pays. L’offre et la demande de stupéfiants explosent simultanément, mettant en péril nos territoires, la santé de nos compatriotes. Qui plus est, ce trafic gangrène déjà nos institutions. En tant que sénateur de la Seine Maritime, je suis particulièrement bien placé pour mesurer l’ampleur de ce « tsunami blanc », qui submerge fortement le port du Havre et inonde ensuite tout le territoire national. Ce mois ci, on y a encore enregistré une saisie record de plus de 2 tonnes de cocaïne, évaluée à 130 millions d’euros. Au delà de ces chiffres impressionnants, ce sont nos forces de l’ordre, douaniers, magistrats, mais aussi élus locaux, qui luttent à armes inégales contre des organisations violentes et déterminées. Nos dockers, et pas seulement eux, se retrouvent pris dans d’infernales spirales d’intimidation, de corruption, de chantage et d’omerta, face à des trafiquants qui rivalisent d’ingéniosité et s’appuient sur une logistique transnationale de plus en plus sophistiquée. De Bogota au Havre, ces routes d’acheminement ont fait du premier port à conteneurs de France une cible privilégiée des narcotrafiquants. Alors que la consommation de cocaïne a presque doublé en un an, cette proposition de loi est une réponse forte et nécessaire à ce fléau. Je tiens à saluer à mon tour la qualité des travaux de nos collègues Étienne Blanc et Jérôme Durain, que ce soit dans le cadre de la commission d’enquête du printemps dernier, à laquelle j’ai pu participer, ou dans l’élaboration des textes Ce texte contient plusieurs mesures attendues. D’abord, le renforcement de l’Office anti stupéfiants et la création du parquet national anti criminalité organisée permettront, je l’espère, une meilleure coordination de la lutte contre ces réseaux.

L’audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Paris a permis aux plus hauts magistrats parisiens de rappeler cette nécessité. Ensuite, dans nos communes, nous savons à quel point certains commerces suspects peuvent être des relais pour le trafic le blanchiment d’argent. Il est indispensable de permettre aux maires de les signaler rapidement et efficacement sur le terrain. Pour autant, il ne s’agit pas non plus de mettre une cible sur le dos de ces derniers ! C’est donc avec sagesse que la commission des lois a supprimé les dispositions conférant aux maires le monopole de l’activation de la mesure. Ils auraient été exposés à un fort risque de représailles, et ce alors même qu’un signalement à l’autorité administrative peut s’effectuer par d’autres moyens. La proposition de loi cible également les recruteurs de jeunes adolescents sur les réseaux sociaux. Ici, nous envoyons un message clair : aucune tolérance pour ceux qui exploitent la jeunesse et compromettent son avenir. Enfin, je salue les dispositions visant à lutter spécifiquement contre la corruption dans les ports et aéroports. Ces infrastructures sont les poumons économiques de notre pays. Il nous faut protéger leurs agents et vaincre l’influence insidieuse des narcotrafiquants sans pour autant – j’insiste sur ce point – risquer de trop ralentir les flux de marchandises. Lors de l’examen de cette proposition de loi en commission, nos deux rapporteurs, Muriel Jourda et Jérôme Durain, ont réalisé un minutieux travail d’adaptation et de sécurisation juridique du texte, qui s’inscrit dans la droite ligne des recommandations formulées par la commission d’enquête. Nous espérons que l’examen en séance de ce texte, si attendu, permettra d’améliorer encore le dispositif. Nous espérons aussi qu’il sera rapidement examiné par l’Assemblée nationale. Mes chers collègues, en adoptant ce texte, nous cherchons à entraver avec détermination ce trafic tentaculaire. Nous protégeons notre jeunesse, défendons nos territoires et réaffirmons que l’État de droit est plus fort que les mafias. Les sénateurs du groupe Union Centriste voteront évidemment en faveur de ce texte. La

nous n’étions que les porte voix de ces nombreuses familles endeuillées, qui désespéraient du manque de réponse de la part de l’État. Personne ne parlait d’elles ni de ces mères qui avaient perdu leur enfant, dealer ou victime innocente, peu importe.

Il nous faudra mettre en place au plus vite le parquet national anti criminalité organisée, qui sera la référence en matière de narcotrafic dans la sphère judiciaire. ailleurs de répondre au besoin de sécurité qu’expriment les citoyens comme les élus, et de soutenir les maires, qui sont réellement démunis face à ce fléau. Il faut mieux protéger les mineurs, bien sûr, les mettre à l’abri des menaces, des violences ou des tortures que leur font subir les trafiquants. J’aurais voulu vous parler également de ces mères célibataires meurtries,

du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Je tiens tout d’abord à saluer le travail remarquable réalisé par Étienne Blanc et Jérôme Durain ; ils ont abouti à deux textes nécessaires et prioritaires pour notre pays.

Le narcotrafic menace au quotidien la sécurité de tous les Français, sur l’ensemble du territoire, en métropole comme en outre mer, dans nos villes comme dans nos campagnes. L’explosion des chiffres ces dernières années

situation concerne surtout nos concitoyens qui n’ont pas d’autre choix que de subir, faute de pouvoir aller vivre ailleurs. Quant aux élus locaux, ils se trouvent en première ligne face aux trafiquants et sont de plus en plus menacés lorsqu’ils leur résistent.

Par ailleurs, ces narcotrafiquants sans état d’âme recrutent aisément des jeunes, des très jeunes, qui sont de plus en plus jeunes. Ces derniers passent des heures, assis sur une chaise, à chouffer et à siffler, et trouvent dans ce trafic l’argent facile qui les conduit systématiquement au décrochage scolaire, à la marginalisation et, parfois, à la mort. Quel gâchis !

Les rapporteurs Muriel Jourda et Jérôme Durain ont souligné l’implication sans faille des services publics chargés de lutter contre ce trafic, mais également l’insuffisance de moyens organisationnels, juridiques et humains dont disposent les acteurs publics.

Bien que ce texte n’y fasse pas référence – on le comprend tout à fait –, n’oublions pas que le narcotrafic pose un véritable problème de santé publique dans notre pays.

Les maires sont aussi les premiers à constater à quel point le trafic de drogue crée une véritable économie parallèle, attirant dans ses filets jusqu’aux plus jeunes. Ils sont encore les premiers à constater comment le narcotrafic déborde sur l’économie de proximité classique : ils voient leurs commerces de quartier ou de village disparaître peu à peu au profit d’autres enseignes, épiceries de nuit comme activités au grand jour, dont chacun sait qu’elles servent en fait de couverture au blanchiment d’argent. C’est ainsi que des rues entières deviennent la propriété et la proie des narcotrafiquants.

le piège du narcotrafic s’est depuis longtemps refermé et qui, désaffiliés, errent dans nos villes et nos villages, le plus souvent dans une très grande précarité, à la recherche de cette dose nécessaire, mais jamais suffisante.

Je vous remercie

Nous nous sommes totalement réorganisés. Ce que nous avons fait contre le terrorisme, il va falloir que nous le fassions contre le narcotrafic, avec, bien entendu, la même détermination dans l’action, la même concentration dans la durée, mais aussi avec un nouvel éventail de mesures, notamment législatives.

Tous les jours, nous voyons ce que la drogue produit : ces vies gâchées, perdues, mutilées ; ces familles otages des mafias, ravagées par ceux qui n’ont aucune pitié pour les enfants, sont par l’appât du gain ; ces quartiers gangrenés malgré tout l’argent public englouti, ces pieds d’immeubles, ces épiceries de nuit, ces commerces bidon. Toutes ces vies volées, toutes ces vies gâchées, ça suffit ! Ce trafic de drogue doit cesser.

Nous devons gagner cette bataille contre les narcotrafics pour préserver notre démocratie et notre État de droit, et pour protéger les plus faibles. La drogue, c’est du malheur et du sang.

la situation actuelle « fait peser un risque grave et insidieux : celui de remises en liberté d’accusés dangereux et, partant, de récidives ». Il en va de même à Marseille, où le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire appellent à un plan Marshall contre le narcotrafic.

Depuis la nuit des temps, dans la mythologie ou même dans la Bible, le banditisme existe. Des cours des miracles à la en passant par les Apaches de la Belle Époque, le crime en bande organisée n’a cessé de se renouveler, toujours guidé par l’appât du gain, sans scrupule ni pitié. Depuis toujours aussi, l’homme tente d’œuvrer pour empêcher que ne s’impose la loi du plus fort, du plus cruel, du plus craint. Pensez aux Tables de la loi : « Tu ne tueras point », « Tu ne voleras point Cette morale judéo chrétienne fonde notre droit. Le pacte républicain, le contrat social et l’acceptation d’une autorité étatique reposent ainsi sur la capacité de l’État à protéger ses concitoyens. L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est clair : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

aux États, il est indispensable de faire face. Il s’agit non plus d’un simple trafic de drogue, mais d’une véritable guerre, déclarée par un ennemi sans aucune limite. Il est donc nécessaire, indispensable et vital de s’armer humainement, techniquement, matériellement et législativement pour doter notre État de droit, notre justice et nos forces de l’ordre des moyens d’éradiquer ce trafic, qui décime notre jeunesse – et pas seulement – et ronge des pans entiers de notre société. tolérance zéro pour les narcos, pour que jamais la loi du crime ne remplace celle de la République

Tous les services de la police judiciaire, tous les offices centraux qui y sont rattachés et tous les organes relevant de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) concourent

Madame la présidente, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, depuis le début de l’après midi, nous nous accordons tous à saluer le travail transpartisan qui a été réalisé. Nous nous accordons tous à constater

un peu trop corporatistes –, qui considèrent qu’il n’y a absolument rien à faire et qui, cet après midi encore, publient des articles et des tribunes affirmant que cette proposition de loi remet en cause les droits de la défense,

je crains fort que nous ne décevions celles et ceux qui attendent que nous prenions notre part de ce combat contre le narcotrafic. Je pense naturellement aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats, aux élus locaux, aux bailleurs sociaux

en 2020, 81 % des 162 204 interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants concernaient uniquement l’usage simple. Autant dire,

À ce titre, l’Ofast, tant par la localisation de son siège que par ses antennes locales, est l’acteur le mieux placé pour orchestrer cette lutte de terrain. Lui confier la coordination des forces de sécurité intérieure sur l’ensemble du territoire garantira un maillage plus efficace et une meilleure collecte de renseignements

à la lumière de l’expérience vécue des élus locaux ruraux, dont je fais partie, d’apporter une réponse pragmatique et opérationnelle à un défi majeur. je vous invite à le soutenir pour mieux protéger nos territoires ruraux et les citoyens qui y vivent. Je me permets d’ajouter, monsieur le ministre, que je ne trouve pas dans l’amendement n° 155 rectifié du Gouvernement cette dimension territoriale rurale.

pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), qui traite des affaires importantes de blanchiment, lesquelles ne sont pas toutes liées au narcotrafic. Quel

aient bien la même longueur ! L’amendement n° 120 de M. Benarroche vise pour sa part à préserver le libre choix des magistrats quant au service d’enquête à saisir. Là encore, cette précision est utile. Nous avons ainsi intégré cette préoccupation, comme en témoigne l’amendement que nous avons déposé en ce sens à

Corinne Narassiguin, pour explication de vote.

lourdement atteinte au principe de finalisation posé par le législateur en 2015, principe selon lequel les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles qui sont prévues à l’article L. 811 3

après avis de la CNCTR. Cette procédure se révèle particulièrement lourde au regard des exigences de réactivité requises par la prévention de la criminalité organisée. Telle est la raison pour laquelle le dispositif initial de la proposition de loi

Afin de donner toute la fluidité requise au fonctionnement de l’autorité judiciaire et de favoriser des échanges sereins entre les différentes juridictions, le présent amendement vise à prévoir la désignation par le procureur de la République, parmi ses substituts, d’un magistrat du parquet faisant office de « référent Jirs

l’action locale, puisque les points de blanchiment peuvent être très territorialisés. Il faut donc que les élus locaux, en coordination avec les services de l’État, aient les moyens de lutter et de proposer des réponses

concrètement contre les actions de blanchiment.

Pour le blanchiment des revenus, un vaste éventail de procédés a été mis en place : la réutilisation directe des fonds criminels, grâce à la réinjection immédiate des espèces dans des secteurs où se pratique le travail dissimulé ; le blanchiment de proximité dans des commerces locaux, souvent ouverts

Il s’agit, par l’intermédiaire du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD ou CISPD), d’associer davantage les élus locaux et l’ensemble des autres acteurs territoriaux dans la lutte contre le narcotrafic, tout en les protégeant individuellement des risques de représailles. Devenus obligatoires dans les communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que dans les communes comprenant une zone urbaine sensible, les CLSPD ou CISPD sont des instances collégiales qui définissent les priorités et les moyens d’action de la commune ou de l’intercommunalité en matière de lutte contre l’insécurité et la délinquance. Or le narcotrafic touche désormais tous les territoires de l’Hexagone comme les outre mer, avec pour corollaire le développement du trafic d’armes et une forte augmentation du narcobanditisme. Face à ce fléau, il faut une réponse forte, coordonnée et partenariale entre la police, la gendarmerie, la justice et les élus. Les maires et les élus des territoires sont d’ailleurs les maillons essentiels du dernier kilomètre du trafic. Ils connaissent la population et les quartiers.

sur le terrain, à commencer par les maires et les policiers municipaux, mais aussi les bailleurs sociaux, à la fois victimes et témoins du petit trafic. Les CLSPD et CISPD peuvent donc se révéler les structures idoines pour mieux coordonner et mieux faire appliquer les mesures de lutte contre le narcotrafic qui figurent dans le présent texte,

Madame la sénatrice, vous souhaitez supprimer la référence à Tracfin au sein de l’article 3 de cette proposition de loi. Celui ci prévoit qu’un groupe thématique local pourra être mis en place afin de traiter des possibilités, pour le maire, de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants en opérant des signalements à Tracfin.

Toutefois, Tracfin, en tant que service de renseignement financier placé sous l’autorité de Bercy, est un acteur essentiel en matière de lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic. Aussi, pour des raisons de cohérence, le Gouvernement émet comme la commission un avis défavorable sur cet amendement. Je

à M. Joshua Hochart. Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des maires en matière de sécurité et d’ordre public, en leur permettant, en concertation avec les représentants de l’État, de prononcer des arrêtés de fermeture administrative d’une durée

recours à des véhicules loués à l’étranger pour leur trafic. La plupart du temps, qu’on le veuille ou non, ces véhicules sont loués dans des agences de location qui elles mêmes savent pertinemment à qui elles les louent et qui sont parfois dirigées par des personnes issues elles mêmes du narcotrafic, notamment dans des pays tels que l’Allemagne et la Pologne. Il suffit de se balader dans les villes de France pour constater que dans nos quartiers, malheureusement, les plaques étrangères pullulent

est à Mme Karine Daniel. Cet amendement vise à inclure les marchands de biens et les promoteurs immobiliers dans la liste des professionnels assujettis aux obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB FT).

Ce rapport souligne en effet que le recours à des structures comme les sociétés civiles immobilières (SCI) pour dissimuler la propriété effective des biens, couplé à la présence de professionnels non soumis au dispositif LCB FT, constitue une vulnérabilité majeure. Le Gafi regrette également que ce risque soit insuffisamment pris en compte dans l’analyse nationale des risques, alors même que certaines autorités rencontrées sur place ont exprimé leur vive préoccupation à ce sujet. L’exclusion des marchands de biens et des promoteurs immobiliers du cadre LCB FT crée une brèche dans notre dispositif de protection contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle affaiblit la traçabilité des flux financiers dans le secteur immobilier, pourtant particulièrement exposé à ces pratiques présent amendement, nous proposons de combler cette faille en soumettant lesdits professionnels aux mêmes obligations que les autres acteurs du secteur. Cette mesure permettra de renforcer la transparence des transactions immobilières, de prévenir les abus et de mieux aligner notre législation sur les recommandations internationales

Quel est l’avis du Gouvernement ? Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Nous prenons toute la mesure de l’exposition du secteur immobilier au risque de blanchiment de capitaux. L’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

les nombreuses enquêtes ouvertes pour blanchiment ou contournement des sanctions économiques montrent que les yachts constituent des vecteurs de blanchiment privilégiés. Il nous semble donc nécessaire de favoriser la vigilance des professionnels concernés par ces transactions en les inscrivant dans la liste des professions assujetties à la LCB FT.

Cela améliorera la traçabilité des transactions et limitera les risques d’utilisation des navires de plaisance à des fins illégales.

Or ces derniers sont en mesure de porter à son attention des suspicions d’intérêt concernant un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général dans le cadre d’une relation professionnelle, que ce soit en tant que salarié, qu’ancien salarié, que membre d’une organisation syndicale représentative du personnel ou encore en tant qu’actionnaire.

état de cause, les sanctions sont à la hauteur des infractions qu’elles pourraient commettre. L’amendement n° 264, présenté par le Gouvernement,

le financement du terrorisme, des personnes soumises aux dispositions de l’article L. 561 2 du code monétaire et financier, conformément aux objectifs de l’article 3 de la proposition de loi. Il est proposé de substituer à l’obligation de certification une obligation de formation professionnelle, soumise au contrôle des autorités de supervision sectorielles mentionnées à l’article L. 561 36 du code monétaire et financier. En effet, ces autorités sectorielles seront les plus à même de s’assurer de la cohérence des dispositifs de formation seront déployés, en fonction des spécificités de chaque profession assujettie : on pense aux risques auxquelles elles sont exposées, ou encore à la maturité des dispositifs internes de lutte contre le blanchiment. En outre, ces autorités sectorielles seraient chargées du contrôle de la bonne mise en œuvre des obligations préventives des professionnels assujettis, y compris de l’obligation

s’appliquent de plein droit dans les collectivités d’outre mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, conformément à leur loi organique, elles doivent être rendues applicables par mention expresse à la collectivité de Wallis et Futuna, régie par une loi ordinaire. Quel est l’avis de la commission ? Je rappelle

La bonne compréhension par ces professionnels des risques auxquels ils sont confrontés dans leurs secteurs respectifs et leur connaissance des obligations qui leur incombent sont des enjeux fondamentaux de la prévention de la criminalité financière. C’est pourquoi nous avons déposé l’amendement que je vous ai présenté à l’instant. faut tenir compte du fait que les situations varient grandement d’un secteur à l’autre. Certains prévoient des formations obligatoires à l’entrée de la profession ; d’autres appliquent des systèmes de formation continue, ce qui rend la certification difficile. certains prévoient l’internalisation des formations au sein des entités ; d’autres, une externalisation. Il convient donc de ne pas défaire ce qui fonctionne actuellement en créant un nouveau dispositif plus complexe, qui échouerait à tenir compte des spécificités de chaque profession.

actuelle, lorsqu’une société française est détenue par une société étrangère, elle n’a aucune obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société mère. Cette lacune prive les administrations françaises et européennes d’une information importante pour identifier les bénéficiaires effectifs réels. Pourtant, ces données sont indispensables pour détecter et démanteler les chaînes de société, notamment extra européennes, mises en place afin d’échapper à l’impôt ou de blanchir des fonds

pragmatique nous semble indispensable pour doter les autorités d’outils adaptés à leurs missions.

ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Cette disposition constitue un outil essentiel de lutte contre les sociétés sans activité réelle, qui interviennent dans les schémas de blanchiment du produit du narcotrafic.

Corinne Narassiguin. Cet amendement vise également à renforcer l’efficacité du mécanisme de régulation des divergences d’information dans le registre des bénéficiaires effectifs. Actuellement, les professions assujetties doivent signaler au greffier du tribunal de commerce toute divergence constatée

de six mois, le greffier puisse procéder à sa radiation d’office. Ce mécanisme renforcerait l’efficacité des signalements en incitant les sociétés à se mettre en conformité dans les délais, tout en maintenant un registre fiable, actualisé et exempt d’entités inactives. Ainsi, cet amendement tend à transformer le signalement de divergences en un véritable levier de régularisation pour les sociétés en activité, tout en contribuant à la fiabilisation du registre pour les entités qui ont cessé leurs activités.

Actuellement, les greffiers des tribunaux de commerce vérifient régulièrement leur registre pour repérer les entités qui n’ont pas rempli leurs obligations de déclaration. Ils envoient alors un courrier, en concertation avec le président du tribunal et le ministère public, pour inviter ces entités à régulariser leur situation dans les plus brefs délais. De nombreuses entités réagissent positivement à cette relance. En revanche, lorsque l’entité ne régularise pas sa situation dans un délai raisonnable alors que le courrier est bien parvenu, le tribunal peut mettre en place la procédure d’injonction prévue par le code monétaire et financier.

: une entité ne pouvant pas être atteinte par les injonctions serait radiée d’office du registre. Cela entraînerait la fermeture des comptes bancaires associés à l’entité, assurant ainsi que seules les entités réellement actives et en conformité figurent dans le registre. Cette mesure renforcerait la fiabilité du RBE et agirait de manière préventive contre les sociétés fantômes, souvent utilisées à des fins frauduleuses.

Quel est l’avis du Gouvernement ? C’est une demande de retrait. En effet, un mécanisme de radiation d’office pour non renseignement des données relatives aux bénéficiaires effectifs ou données erronées est déjà prévu dans cette proposition de loi.

L’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales dispose que « pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale,

amendement vise à permettre aux agents de la police des finances – c’est à dire les agents des douanes et des services fiscaux qui exercent leur mission sous la responsabilité des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires – de disposer d’un accès direct

Cet amendement vise à autoriser les douanes à accéder directement aux données pertinentes contenues dans les traitements des opérateurs de la logistique et du transport portuaire et aéroportuaire.

La menace criminelle pèse sur les plateformes logistiques portuaires et aéroportuaires, ainsi que sur les centres de fret postal et express, et atteint un niveau d’intensité inédit. Dans ces conditions, le présent amendement vise à autoriser les agents des douanes à accéder aux données contenues dans les traitements automatisés des entités des secteurs du transport et de la logistique, ainsi qu’à les exploiter, notamment au travers d’analyses de risques, afin de renforcer la capacité de détection. Il convient de donner aux douanes les moyens de faire face aux nouvelles formes de criminalité et aux mutations des circuits de fraude, qui empruntent désormais majoritairement les circuits commerciaux et logistiques légaux.